Monsieur le président, La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Arnaud de Belenet.

Enfin, je ferai le point sur quelques sujets sur lesquels il ne me semble pas impossible de converger ; je m'en remets avec confiance à l'intelligence collective dont le Sénat est capable.

près d'une cinquantaine de réunions ont été organisées en 2018 et au début de 2019 avec les neuf organisations syndicales de la fonction publique et les représentants des collectivités locales et des employeurs hospitaliers. Vous disiez avoir également rencontré, dans un esprit

L'ambition de ce texte est d'adapter les règles applicables aux 5,5 millions d'agents du service public. Cela n'a rien d'une mince affaire ; c'est même de l'orfèvrerie, en particulier en France, où la fonction publique est associée, organiquement, à une certaine idée de la Nation.

Comment, alors, ne pas accueillir avec quelques motifs de satisfaction un texte qui met en oeuvre les outils indispensables à la révision opérationnelle de la fonction publique, sans préjudice des lois statutaires de 1946 et de 1983 ? la méthode, j'ai évoqué les 5,5 millions d'agents du service public. Ce n'est pas qu'un luxe de précaution sémantique. En effet, à l'heure où l'on se plaît à compartimenter la fonction publique en corps, en cadres d'emploi, en emplois fonctionnels, que sais-je encore ?, le titre V du présent projet de loi, consacré à l'égalité professionnelle, a ceci d'opportun qu'il nous rappelle une chose essentielle : il faut à tout prix cesser de voir des catégories statutaires là où l'on trouve d'abord des serviteurs de la Nation qui méritent, chaque jour, d'être salués et encouragés.

de vue, le Gouvernement n'est pas en peine. C'est vrai, en premier lieu, pour les services publics et leur adaptation aux attentes des usagers ; l'une des dernières avancées notables consiste en l'instauration d'un droit à l'erreur,

d'adapter et de renforcer le dialogue social dans la fonction publique, que l'on peut parfois qualifier d'atone, en proposant une réforme des organes de proximité : les futurs comités sociaux pourront trancher l'ensemble des questions liées à la gestion des ressources humaines.

nationale, a indiscutablement su se saisir d'enjeux majeurs pour les agents de la fonction publique. Notre commission s'est efforcée de renforcer les souplesses offertes aux employeurs territoriaux, notamment en élargissant le recours aux agents contractuels, en encourageant les recrutements sur titres pour des agents disposant déjà d'un diplôme d'État. Je salue, notamment sur ce point, le rapport

Enfin, la commission des lois a opportunément garanti de nouveaux droits aux agents publics en les rendant éligibles au congé de proche aidant et en prévoyant que les fonctionnaires de genre féminin disposeront d'une heure par jour pour allaiter leur enfant, comme dans le secteur privé. Le Sénat a ainsi participé, au travers des

parfois, peut-être, de posture, ne gâchent pas, non pas cet échange d'amabilités, mais cette véritable contribution au sujet majeur qu'est la transformation de notre fonction publique.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je concentrerai mon propos sur les conséquences de ce projet de loi sur la fonction publique hospitalière. Dans cet esprit, je regrette que, du fait de l'inflation législative, la commission des affaires sociales n'ait pu se saisir pour avis de ce texte, comme je l'avais proposé. Alors que les hôpitaux connaissent une crise majeure, que leur personnel est au bord de l'explosion, que les agents multiplient les actions, depuis des mois, pour dénoncer leurs conditions de travail et la dégradation de la prise en charge des patients,

Vous proposez, à l'article 28, une externalisation des missions des personnels, mais avez-vous entendu des soignants, des agents administratifs, ou encore des ouvriers qui travaillent dans les établissements publics de santé vous en faire la demande ?

fonctionnaires d'évoluer tout au long de leur activité professionnelle. Votre obsession de vouloir casser le statut des fonctionnaires, que vous dénoncez comme d'affreux privilégiés tandis que vous épargnez les tenants du CAC 40, est tout simplement indécente pour ces hommes et ces femmes qui nous soignent ! Vous étendez au secteur public les réformes appliquées au secteur privé depuis les ordonnances Macron ou la loi El Khomri, en réduisant à peau de chagrin les instances représentatives du personnel, pour tuer toute concertation. Ainsi, vous ne trouvez pas mieux que de supprimer les CHSCT, Comment le comité social d'administration, instance fourre-tout censée les remplacer, interviendra-t-il quand des agents menaceront de sauter par la fenêtre parce qu'ils n'en peuvent plus ? On en est bien là aujourd'hui, mes chers collègues, tant les restrictions budgétaires faites sur le dos des hôpitaux depuis des années entraînent une perte de sens, un épuisement des personnels et une profonde souffrance au travail. Comment cette instance pourra-t-elle mener des actions de lutte contre les violences sexistes et le harcèlement ? Cela m'amène à aborder, pour conclure, le volet de ce texte Comme l'a souligné Éliane Assassi, les quelques mesures proposées sont loin d'être suffisantes. Une fois de plus, la grande cause nationale de ce quinquennat mobilise bien peu votre gouvernement, monsieur le secrétaire d'État ! Le statut de la fonction publique est un outil vivant que l'on se doit d'améliorer au fil du temps pour mieux servir l'intérêt commun, mais vous faites le contraire : vous le détruisez et vous allez amplifier la crise dans la fonction publique hospitalière. Voilà une raison supplémentaire pour voter contre ce projet de loi, qui, en mettant à mal les trois principes fondateurs de la fonction publique, aggravera les conditions de travail des fonctionnaires, dégradera les services rendus à la population

Leur mission fondamentale est de permettre à tous nos concitoyens d'accéder à un patrimoine commun, le service public, leur ouvrant le droit à la santé, à la sécurité, à l'éducation, à la culture, à la mobilité, à la justice et à tout ce qui concourt à notre vie collective. Le service public, ne l'oublions pas, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, le bien commun de la Nation. La fonction publique est en souffrance, non parce qu'il y aurait trop de fonctionnaires, mais parce qu'ils ne sont pas toujours là où il le faudrait, du fait de choix dictés par des impératifs budgétaires réalisés à leurs dépens et à ceux des usagers. Comment, à l'heure où nous engageons l'examen de ce texte, ne pas penser au personnel hospitalier et, en particulier, à celui des urgences, au personnel pénitentiaire, victime de prises d'otages, aux agents de la force publique, éreintés par la crise des gilets jaunes,

Aujourd'hui, nous tenons, avant toute autre chose, à apporter tout notre soutien à l'ensemble de la fonction publique et de ses agents, dont nous saluons le professionnalisme, l'intégrité et le dévouement. C'est ce soutien qui guidera nos positions et nos interventions tout au long de nos débats. La force de notre fonction publique est le statut des fonctionnaires, qui oblige et protège ses agents. Permettez-moi de faire un rappel rapide, mais nécessaire. La fonction publique est consubstantielle de la République. Son statut n'est pas un héritage désuet du XX siècle ; c'est une opportunité. Constitué d'un ensemble de droits et de devoirs, le statut est un cadre qui a su se moderniser, de sa création, en 1946, aux quatre lois de 1983, 1984 et 1986, qui forment aujourd'hui le statut général des fonctionnaires. Il repose sur trois principes, qui restent modernes. Le premier, c'est l'égalité. L'entrée dans la fonction publique se fait par la voie du concours, qui garantit l'égal accès aux emplois publics et la sélection par la compétence. Le concours est le meilleur rempart contre le copinage, le favoritisme et le clientélisme. Le deuxième, c'est l'indépendance. Les fonctionnaires doivent être protégés de la conjoncture et de l'arbitraire politiques. La fonction publique française repose donc sur le système de la carrière, où le grade est distinct de l'emploi. Servir l'État, ce n'est pas servir une société privée : c'est une fonction sociale, qui s'apprécie sur une longue période aménagée à cet effet en carrière. Le troisième, c'est la citoyenneté. Les fonctionnaires disposent des mêmes droits que les autres citoyens- liberté d'opinion, droit syndical et droit de grève, pour prendre les plus emblématiques -, mais ces droits doivent être conciliés avec des obligations propres à la fonction publique en matière de neutralité, de déontologie, de laïcité, de discrétion et d'information du public. Autant de principes qui sont aujourd'hui menacés par ce projet de loi. En effet, monsieur le secrétaire d'État, avec cette réforme, si vous ne vous attaquez pas frontalement au statut, vous le contournez. Vous élargissez massivement les possibilités de recruter des agents contractuels en lieu et place des fonctionnaires, mettant en concurrence les seconds avec les premiers. Vous multipliez ainsi les risques d'emplois de complaisance, au détriment de la compétence, et vous réduisez fortement les perspectives de carrière des fonctionnaires qui ont fait le choix de s'engager en faveur de l'intérêt général. De plus, vous renforcez la précarité des agents publics, à l'image du nouveau contrat de projet, ou encore du détachement d'office auprès d'opérateurs privés en cas d'externalisation de services ou de missions. En revanche, vous restez silencieux sur la reconnaissance de l'engagement de nos concitoyens au sein de la fonction publique et sur les possibilités d'évolutions professionnelles, notamment par le biais de la formation continue, tout au long de leur carrière, ou de congés de conversion. Ainsi, en ouvrant très largement le recours au contrat, vous faites le choix de la banalisation de la fonction publique et de l'exercice de l'État ; vous faites le choix,, de l'affaiblissement de l'action publique. Votre projet de loi remet en cause de manière inédite le dialogue social à tous les étages de la fonction publique. D'une part, il fusionne des instances, au détriment de celles qui sont compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, alors même que la santé au travail est un enjeu primordial dans un contexte de restructurations annoncées. D'autre part, il réduit les attributions des commissions administratives paritaires, qui sont aujourd'hui consultées sur toutes les décisions individuelles. Vous nous dites que ces instances sont source de rigidité, alors qu'elles n'ont aucun pouvoir décisionnel, qu'elles garantissent la transparence des décisions et qu'elles permettent souvent de renforcer l'acceptabilité des décisions auprès des agents.

vous avez négligé les organisations syndicales, en ne tenant pas votre engagement, plusieurs fois répété, de publier les projets de décrets en même temps que le projet de loi. Rappelons que ce texte, que vous dites attendu de tous, fruit d'une prétendue concertation intense, a fait l'objet d'un rejet unanime de la part des neuf organisations syndicales de la fonction publique. Vous ne respectez pas plus les parlementaires en utilisant, une fois de plus, la procédure accélérée et en recourant massivement aux ordonnances. En résumé, ce projet de loi n'est rien d'autre qu'une volonté de dégradation organisée des services publics ; il contribue à la stigmatisation de ceux qui les mettent en oeuvre. Il ne résoudra ni les problèmes de fonctionnement de nos services publics ni le malaise de nombreux agents. Il ne répondra pas plus aux demandes des citoyens désireux de plus de proximité. La majorité sénatoriale présente ce projet de loi comme une boîte à outils.

il dessine en creux la conception que le Gouvernement se fait du service public et de l'État. Penser la fonction publique, c'est penser l'action publique dans notre société. Pour nous, son histoire est républicaine. Elle a une place singulière dans l'organisation sociale et politique du pays. Elle contribue à l'émancipation individuelle des Français. Elle est le bras armé des libertés publiques, de la solidarité, de la fraternité républicaine et de la laïcité ; bref, de l'intérêt général. Ce texte est malheureusement un projet d'affaiblissement du service public, qui prépare la mise en oeuvre du plan Action publique 2022 et la suppression de 120 000 emplois.

le projet de loi de transformation de la fonction publique aborde une réforme capitale, dont nous attendons qu'elle permette à l'État de se doter des instruments législatifs nécessaires pour la redéfinition de l'action publique, tant à l'échelon national que dans nos territoires, afin de se recentrer sur les services jugés utiles par nos concitoyens. Les récents mouvements sociaux traduisent le décalage qui s'est creusé depuis des décennies entre les usagers et leurs services publics, qu'ils jugent inadaptés ou trop éloignés. Au sein des fonctions publiques, les crises se multiplient crise de vocation dans les juridictions et les écoles, crise de l'épuisement dans les hôpitaux, les casernes, les prisons et les commissariats, crises de nerfs aux finances. Ce décalage entre, d'un côté, des administrés insatisfaits et, de l'autre, des agents épuisés doit nous conduire, sur toutes les travées de cet hémicycle, à aborder avec lucidité, plutôt qu'avec idéologie, la question de la réaffectation des moyens administratifs humains par service et par zone géographique, en fonction des besoins exprimés sur le terrain et dans le cadre d'une dépense publique maîtrisée. À force de temporisations, la situation s'est cristallisée : il y a désormais urgence à agir. Le premier obstacle à la réforme de l'État réside dans l'importance du nombre d'agents publics. On ne transforme pas une organisation rassemblant 5,5 millions de personnes comme une entreprise de plusieurs dizaines de salariés. Mais là où d'autres grandes démocraties sont parvenues à faire leur administratif- je pense par exemple

et de la fonction publique, dès la circulaire du 23 février 1989. On peut également considérer que certaines positions syndicales conservatrices ont eu leur part de responsabilité dans les difficultés d'adaptation des services : alors qu'il aurait fallu saluer et encourager l'ouverture de l'emploi public à des profils issus du privé, le recours aux nouvelles technologies, ces éléments ont été systématiquement perçus comme des attaques portées au statut. Ainsi, dans bien des administrations, la transition numérique s'est fait dos au mur ou en catimini, avec la suppression des fonctions de secrétariat. Les nouvelles générations de fonctionnaires en paient aujourd'hui le prix fort.

Plusieurs nouveaux outils que vous proposez devraient permettre le redéploiement d'agents publics là où ils seront utiles : je pense aux instruments d'encouragement à la mobilité géographique et à l'intérieur de la fonction publique, prévus à l'article 26, ou encore au détachement d'office, qui devrait faciliter les externalisations et permettre aux décideurs publics de tester différentes formes de gestion d'un service public. Vous vous attaquez également à la crise des vocations en offrant aux fonctionnaires en souffrance une voie facilitée de reconversion professionnelle hors du secteur public par la consécration d'une forme de rupture conventionnelle et par l'ouverture du recours à la forme contractuelle entre les employeurs publics et les agents. Il s'agit d'une adaptation intelligente aux aspirations de mobilité professionnelle des « enfants du numérique », comme les nommait le philosophe Michel Serres il y a peu encore. Cependant, nous y mettons plusieurs conditions. Il est d'abord nécessaire que, comme en matière de concours, l'accès à l'emploi public par voie contractuelle offre des garanties de transparence et d'équité satisfaisantes. Il est question pour nous de passer non pas à un, mais à un système de recrutement hybride destiné à permettre le recrutement de profils plus variés pour enrichir l'action publique. L'apport de ces agents contractuels doit être mieux valorisé, afin qu'ils ne soient pas traités comme de simples variables d'ajustement, moins rémunérés et moins protégés que les agents statutaires. C'est le sens de plusieurs de nos amendements relatifs au contrat de projet, à la requalification en CDI, ou encore à la reconnaissance de l'expérience de ces personnels au moment de leur recrutement ou, par la suite, lorsqu'ils se décident à passer des concours.

cela ne devrait pas être le cas s'ils étaient rémunérés dans des conditions identiques. On est donc loin d'un développement de la contractualisation dans des conditions égales entre fonctionnaires et contractuels nous sommes particulièrement vigilants à ce que les allers-retours entre le secteur public et le secteur privé se fassent dans des conditions plus satisfaisantes pour l'intérêt général. Plusieurs travaux parlementaires ont mis en lumière les défauts du système de contrôle déontologique actuel.

Pour clore ce sujet, les fonctionnaires doivent envisager l'augmentation du nombre d'agents contractuels non comme la remise en cause de leur statut, mais comme l'enrichissement d'un corps administratif unique par une nouvelle composante destinée à pallier les défauts de la composante historique, laquelle n'a pas vocation à disparaître. Je crois que cette approche pragmatique est également partagée par nos deux rapporteurs, dont je tiens à saluer le travail considérable. À quelques réserves près, nous soutenons les modifications apportées au texte telles que le meilleur encadrement des habilitations à légiférer par ordonnances, la suppression de l'habilitation réformant le dialogue social qui n'a pas été assez préparée, le maintien des questions de rémunération et d'avancement dans le champ de compétence des CAP, et les modifications introduites en faveur des employeurs publics locaux qui leur offrent ainsi de plus grandes marges de manoeuvre dans la gestion des ressources humaines. Nous proposons d'ailleurs de renforcer le droit de regard des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre des détachements d'office de fonctionnaires d'État lorsqu'ils auraient des répercussions locales, comme le dénoncent déjà les Sur d'autres points, comme la suppression de la prime de précarité pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière, nous sommes nettement plus circonspects. Cela dit, si nous soutenons le développement de la politique du handicap au sein de la fonction publique nous avons entendu l'argument du Gouvernement, qui souhaite faire converger les normes publiques et privées en la matière, nous ne partageons pas votre conviction, monsieur le secrétaire d'État. De la même manière, nous espérons que nos échanges pourront apporter une solution à l'épineuse question du financement de l'apprentissage. Je conclurai en exprimant quelques regrets sur un outil de management qui me paraît insuffisamment encouragé par le texte : celui de la valorisation du mérite par l'individualisation des primes. On connaît l'attachement des syndicats aux primes d'intéressement collectif, qui sont particulièrement justifiées dans des services sous tension. Le projet de loi prévoit justement de les étendre aux services hospitaliers. Pour autant, dans de grands organigrammes comme ceux des ministères, nous considérons que de nouveaux outils auraient pu être mis en place pour distinguer le mérite individuel dans la construction de la carrière. Certes, quelques initiatives ont été développées avec des partenaires, comme les Victoires des Acteurs publics. Le remplacement de la notation par un entretien individuel va aussi dans le bon sens, mais les liens entre promotion et mérite pourraient être davantage renforcés, quand bien même cela atténuerait le sacro-saint principe de l'ancienneté.

en propos liminaire, je rappelle que ce sont 5,5 millions d'agents qui oeuvrent au quotidien pour la bonne organisation des services publics. Je souhaite saluer leur travail à cette tribune. La fonction publique constitue notre bien commun. Il convient de la préserver tout en modernisant son organisation. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, bien qu'il ne traduise pas une réelle vision de l'action publique, comporte une palette d'outils pouvant permettre une meilleure gestion des ressources humaines. humaines. Il ne procède pas à une véritable « transformation » de la fonction publique, mais il comporte une série de modifications, souvent techniques, dans trois domaines : la simplification du dialogue social et les nouveaux outils managériaux l'élargissement du recours aux contractuels ; le renforcement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il vise également à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur des thèmes sensibles : le dialogue social, la formation des agents, ce qui comprendrait la réforme de la haute fonction publique, et la santé au travail. Je me réjouis que le travail en commission ait notamment eu pour objectif de préserver les spécificités de la fonction publique territoriale et de mieux répondre aux attentes des employeurs locaux. En effet, la fonction publique territoriale constitue un maillon indispensable de l'organisation décentralisée de la République, notamment pour la gestion des services publics de proximité, comme les polices municipales, les cantines et les crèches. Je me réjouis que la commission ait donc donné plus de prévisibilité aux élus locaux en obligeant l'État à publier une feuille de route triennale dans laquelle il indiquerait l'incidence financière sur les budgets locaux de ses décisions en matière de ressources humaines. Je me félicite Je me félicite également de ce que la commission ait veillé à accorder davantage de souplesse, notamment en permettant aux communes de moins de 2 000 habitants de pourvoir l'ensemble de leurs emplois par voie contractuelle et en élargissant le contrat de projet aux agents de catégorie C. Par ailleurs, je tiens à souligner la volonté de la commission de donner de nouveaux outils aux employeurs territoriaux en limitant à cinq ans la durée de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, en facilitant le licenciement pour insuffisance professionnelle et en renforçant le régime disciplinaire, tout en réaffirmant le caractère paritaire des conseils de discipline. Enfin, je suis satisfait que la commission ait sécurisé le financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale. La fonction publique territoriale emploie actuellement 14 000 apprentis. Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les régions ne sont plus compétentes pour financer les centres de formation des apprentis.

Or cette somme paraît bien trop élevée au regard du budget du CNFPT et risque de remettre en cause les formations dispensées aux autres agents territoriaux. Dans un souci de compromis, la commission a proposé que tous les acteurs s'engagent pour soutenir l'apprentissage dans les collectivités territoriales en prévoyant que 30 % des coûts de formation soient pris en charge par l'État et 20 % par le CNFPT. Avant de conclure, je souhaite saluer le considérable travail fourni par les rapporteurs sur ce texte très technique et dont le champ est large. Je souhaite également vous faire part de mon regret concernant le choix du Gouvernement d'engager la procédure accélérée sur ce projet de loi essentiel pour la fonction publique. Ah oui ! Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'examen en commission a permis d'élargir la palette d'outils pouvant permettre une meilleure gestion des ressources humaines tout en respectant les droits des agents publics et les grands principes du statut général.

apparaît en décalage avec l'ambition de l'intitulé. Tel est encore le cas avec ce projet de loi de transformation de la fonction publique qui traduit davantage un assouplissement et une adaptation de la fonction publique qu'une véritable transformation. Nous ne sommes pas véritablement ici dans la rupture ! Ah non ! Néanmoins, nous approuvons la volonté de l'exécutif de faire évoluer l'environnement, l'environnement, les métiers et les missions des agents publics, afin de les adapter aux défis de notre temps. Les membres du groupe Union Centriste ne sont pas dans l'immobilisme. dans le centrisme ... Ils admettent bien volontiers que, s'il a sa raison d'être, le statut de la fonction publique ne saurait être figé. Nul ne peut sérieusement le contester : l'apparition de nouveaux métiers commande de nouvelles compétences. D'ailleurs, les agents du service public eux-mêmes réclament de nouvelles mobilités dans le temps et dans l'espace. En revanche, nous regrettons que le texte- tout du moins dans sa version initiale -s'arrête au milieu du gué. Il confine, hélas !, trop souvent au salmigondis de mesures disparates, se contentant d'empiler des dispositifs techniques, arides, desquels ne découle aucune philosophie d'ensemble. L'occasion est pour ainsi dire manquée de réformer en profondeur la fonction publique et de fixer, pour elle et pour les 5,5 millions d'agents qui l'animent au quotidien, un authentique cap vers l'avenir. Car si les trois versants de la fonction publique recouvrent des missions très différentes, qui relèvent de corps, de cadres d'emploi et de métiers eux-mêmes multiples, tous ont en commun une même finalité : la grandeur du service public. sujet ô combien décisif, aux ramifications multiples, comme ont tenu à nous le rappeler les Français à l'occasion du grand débat L'attente de nos concitoyens à l'égard du service public est immense d'un bout à l'autre du territoire. Elle est à la hauteur de ce qu'il représente dans notre pays en termes de service rendu, d'emploi et de cohésion sociale. Nous avons conscience de la complexité du défi qui nous est posé : d'un côté, nos concitoyens réclament une plus large intervention de l'État et un retour à des services publics de proximité plus poussés ; de l'autre, ils guettent « sourcilleusement » le niveau de pression fiscale. Il était donc devenu indispensable d'agir. À cet égard, nous ne pouvons que nous féliciter de l'action engagée par le Gouvernement. Sans doute les objectifs ne sont-ils pas toujours clairs, faute d'avoir été nettement exposés par le Gouvernement lui-même. Là réside en partie, je crois, l'explication à l'opposition de l'ensemble des organisations syndicales. L'avenir du secteur public aurait dû en effet susciter un plus vaste débat, afin que soit discuté l'ensemble des questions afférentes à la carrière des fonctionnaires, au statut au statut de la fonction publique et à son avenir, à la rémunération, à la retraite, de façon à pouvoir apporter, en toute transparence, des réponses d'ensemble aux agents publics, ainsi qu'à nos concitoyens. L'enrichissement du texte avant même l'issue de la première lecture est très parlant. Il est révélateur en tout cas des imperfections et incohérences de départ.

Je tiens, à cet égard, à saluer le travail remarquable accompli par les deux rapporteurs, Catherine Di Folco et Loïc Hervé, qui ont abordé sans dogmatisme aucun ... Aucun dogmatisme, attitude toujours constructive les différents volets de ce projet de loi, qu'il s'agisse des instances de dialogue social, de l'élargissement du recours aux contractuels, de la réforme du cadre déontologique

leur initiative ou sur l'initiative de certains de nos autres collègues, ont permis d'améliorer substantiellement le texte transmis au Sénat par l'Assemblée nationale. L'obligation pour l'État de présenter une feuille de route triennale indiquant tout à la fois ses orientations en matière de rémunération, de déroulement de carrière, de formation et de mobilité des agents publics participe ainsi, et de manière transversale, au besoin et de manière transversale, au besoin de visibilité que réclament nombre d'élus partout dans nos provinces. J'espère que l'article 2 prospérera à l'issue de l'examen du texte par la Haute Assemblée. De même, la modification de la périodicité du rapport social unique, qui deviendrait biennal plutôt qu'annuel, ménage davantage de souplesse

que les vider de leurs compétences, ainsi que vous le proposez, n'améliorerait en rien le dialogue social au sein de la fonction publique. Eh en supprimant leurs compétences, vous créerez des rapports conflictuels, eux-mêmes source de défiance, au détriment finalement de l'efficacité du service public. Soyez attentif aux arguments du Sénat et à sa sagesse habituelle en ne rayant pas d'un trait de plume la compétence des CAP en matière d'avancement et de promotion. Je me réjouis surtout des nombreux apports de la commission allant dans le sens d'une plus grande souplesse offerte aux employeurs locaux. S'agissant de l'élargissement du recours aux contractuels, point clé de ce projet de loi, quel meilleur garant du principe d'égal accès aux emplois publics que les autorités locales elles-mêmes ? Là encore, la réécriture de l'article 6 par la commission des lois du Sénat me semble salutaire en ce sens qu'elle garantit l'adaptation des recrutements aux besoins des collectivités locales.

que vous rejoignez la position de la chambre haute, et veillerez à ne pas attenter à la libre administration des collectivités en ne faisant pas s'immiscer l'État dans les relations entre exécutifs locaux et directeur général des services. Très bien ! De même, je ne doute pas que vous rejoindrez notre proposition et étendrez à tout type d'emploi le recours au nouveau contrat de projet, sans exclusion des emplois de catégorie C. Au titre des lacunes originelles du texte, le Gouvernement a oublié deux points majeurs au sujet du recrutement, seulement traité sous l'angle des contractuels : je veux parler de l'apprentissage et des concours. J'aimerais d'abord dire un mot sur le développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales, point central du dynamisme économique de nos communes, de nos départements et de nos régions. Notre cher collègue Loïc Hervé l'a rappelé : les quelque 14 000 apprentis du secteur public sont les grands oubliés de la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La nouvelle mouture de l'article 22 B du présent projet de loi y remédie en proposant notamment d'associer l'État au soutien et au financement de l'apprentissage dans les collectivités par le truchement d'un prélèvement sur recettes. bon coeur ! Il s'agirait là d'un investissement d'avenir, non d'une politique hasardeuse et dispendieuse ! J'aimerais ensuite saluer, au travers du nouvel article 33 , d'emplois des concours sur titres, aujourd'hui réservés aux seules filières sociales, médico-sociale et médico-technique. J'espère vivement que ces deux apports du Sénat recevront toute l'attention qu'ils méritent de la part du Gouvernement. Je le soulignais en préambule, il est difficile de décortiquer ce projet de loi mesure par mesure, preuve qu'il manque de cohérence globale S'agissant de la déontologie, de la transparence et de l'égalité entre les femmes et les hommes, nous sommes bien sûr très favorables aux mesures contenues dans le texte, ainsi qu'aux nouvelles avancées obtenues en commission. Cela a été rappelé, le Gouvernement a eu le grand mérite d'intégrer à son projet de loi plusieurs propositions du Sénat, en particulier l'harmonisation du temps de travail et l'introduction de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Il serait bien inspiré de poursuivre dans et de conserver l'ensemble des préconisations du rapport de nos collègues Catherine Di Folco et Didier Marie, lesquelles visent à maints égards à renforcer l'intégration des agents en situation de handicap.

L'extension du congé de proche aidant aux agents publics, d'une part, la possibilité pour les femmes salariées de la fonction publique d'allaiter leur enfant pendant leur temps de travail, d'autre part, sont deux mesures sociales garantissant l'équité entre les entre les secteurs public et privé. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste est favorable à l'esprit de ce texte, quelles que puissent en être par ailleurs les insuffisances. Nous voterons bien entendu en faveur de ce en espérant que les recommandations et améliorations du Sénat trouveront un écho auprès du Gouvernement et de nos homologues députés. Nombre d'entre elles sont attendues avec impatience par nos agents publics, nos concitoyens et nos territoires

des dispositions concrètes proposées par ce gouvernement pour réformer les moyens de l'action publique. J'avoue que nous étions fort impatients d'apprendre ce qui suivrait les déclarations du président Macron, qui nous avait promis un choc d'efficacité concernant les effectifs de l'État d'ici au terme du quinquennat. Car nous étions restés sur notre faim après les conclusions du comité Action publique 2022, dont les traductions concrètes tiennent finalement moins du big-bang annoncé que du feu de Bengale. Nous retenions donc notre souffle dans l'attente de ladite transformation de la fonction publique ! Mais comme l'ont très bien relevé les rapporteurs, Catherine Di Folco et Loïc Hervé, pour se hisser à la hauteur d'une telle ambition, il manquait à ce projet de loi

des besoins de la fonction publique plus efficace et les évolutions de carrières plus stimulantes. On ne peut que les saluer. Ces avancées sont d'autant plus salutaires aux yeux des sénateurs de mon groupe que certaines dispositions emblématiques avaient été proposées par le Sénat, comme l'harmonisation par le haut du temps de travail annuel des agents ou la possibilité de procéder à des ruptures conventionnelles dans la fonction publique. Ces deux mesures incarnent la double nécessité qui doit guider tout employeur public : d'un côté, la gestion rigoureuse des moyens publics ; de l'autre, la souplesse au service de l'efficacité. Cette équation est plus facile à poser qu'à résoudre, et les élus locaux connaissent le difficile équilibre entre un service exigeant pour la population, qui sera effectué par des agents qui s'épanouissent dans leur métier, et des perspectives professionnelles renouvelées. Je veux donc saluer les deux rapporteurs de la commission des lois pour avoir mené cet exercice d'équilibre au bénéfice d'un texte enrichi en ayant su relever les trois défis qu'ils s'étaient mieux répondre aux besoins exprimés par les collectivités locales, davantage gratifier la qualité du service des agents et donner enfin sa place au handicap. Je tiens particulièrement à remercier Catherine Di Folco des nombreuses dispositions qu'elle a intégrées au texte du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi en commission, et qui touchent à la fonction publique territoriale. Elle a su créer des outils efficaces pour répondre aux attentes que les élus locaux ont fait remonter en participant massivement à la consultation lancée auprès d'eux par le Sénat. Parmi celles-ci, je saluerai la limitation à cinq ans de la durée maximale de prise en charge des agents placés dans la catégorie des fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Cette mesure met un terme à des situations invraisemblables : certains fonctionnaires, sans occuper de poste, étaient pris en charge depuis plus de vingt ans par les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale. Comment, mes chers collègues, peut-on regarder ses administrés dans les yeux et leur dire qu'on ne peut recruter tel ou tel agent utile pour la petite enfance, le sport ou la culture quand perdurent de telles situations ? Quelle image donne-t-on aux agents de leur statut, censé être tourné vers le service de la collectivité, quand celle-ci n'est pas capable de mettre à profit leur énergie et leurs compétences ? Quant à l'amendement déposé par François Bonhomme et massivement soutenu par le groupe Les Républicains, il va dans le même sens, en rationalisant les conditions de liquidation de la retraite d'un fonctionnaire momentanément privé d'emploi. Au sein de la fonction publique territoriale et particulièrement dans les communes, il existe un lien affectif entre les agents et la collectivité qu'ils servent. Voilà pourquoi l'implication de ces personnels doit être récompensée à hauteur de leurs mérites. C'est même là une demande formulée par les élus locaux eux-mêmes, qui est massivement apparue dans la consultation menée par le Sénat. C'est pourquoi je salue l'idée des rapporteurs de rapprocher l'évaluation de la performance aux résultats du service tout entier, ce qui a vocation à affermir le lien entre les agents d'une même équipe dont les efforts tendent vers un objectif commun. L'un des aspects qui me paraît primordial dans ce texte est la prise en considération des spécificités territoriales qui vise à favoriser l'installation des fonctionnaires territoriaux dans les zones rurales ou enclavées. mesure représente une avancée importante, voire essentielle, qui peut constituer un pacte gagnant pour les collectivités et les agents eux-mêmes. Un mot sur ce point, monsieur le secrétaire nous avons en partage d'être issus du même territoire à profil plutôt rural. Les agents qui permettent d'y faire perdurer la présence de l'action publique ne représentent jamais des dépenses superflues. La diminution des services publics de proximité n'est pas pour rien dans le sentiment d'abandon qui s'est manifesté si fortement depuis le déclenchement du mouvement des gilets jaunes, ou lors de bon nombre de scrutins depuis une dizaine d'années. Il faudra s'en souvenir lorsque le gouvernement que vous représentez proposera un nouvel acte de la décentralisation avec à la clé, espérons-le, des moyens humains mieux répartis au coeur des territoires. Dans l'immédiat, nous serons vigilants, et je ne vous cache pas notre inquiétude quant au redéploiement de certains services, comme ceux du Trésor public. Plus de reconnaissance, un dialogue social modernisé et de meilleures perspectives de carrière permettent de remettre les agents au centre de l'action publique. Cette place restaurée et cette confiance réaffirmée doivent aller de pair avec un esprit de responsabilité réactualisé. Il y va tout simplement de l'image des 5,5 millions d'agents publics. Je salue donc, monsieur le secrétaire d'État, le pragmatisme dont vous avez fait preuve en reprenant les propositions du Sénat concernant l'harmonisation du temps de travail. Vous proposez ainsi de mettre un terme aux dérogations au temps de travail annuel qui ne se justifiaient que par des pratiques locales, certes légales, mais que nos concitoyens, lesquels sont aussi, par le biais de leurs élus, les employeurs, ne comprennent plus. du groupe Les Républicains a décidé de soutenir l'initiative de nos collègues Christine Lavarde et Dominique Estrosi Sassone : elles nous ont alertés sur le phénomène des grèves perlées, qui créent un rapport de force parfois déséquilibré entre les grévistes cessant leur activité en roulement et le service, qui peut être saturé et perturbé. Dans le cadre d'un conflit social, le mouvement de grève conserverait

ne l'est pas assez dans certaines zones, nous savons qu'elle est enviée pour sa fonction publique dévouée, compétente, honnête et efficace. à cette dernière que de déployer pleinement son potentiel en se modernisant et en traçant de nouvelles voies plus enthousiasmantes pour nos agents. Si ce texte comporte de bons outils, il a besoin du savoir-faire du Sénat pour parachever son oeuvre : voir éclore une fonction publique plus pragmatique, au service des citoyens de l'ensemble de nos territoires. La parole

Mme Céline Brulin. Monsieur le secrétaire d'État, alors que le Président de la République avait vaguement laissé supposer le possible abandon de la suppression de 120 000 postes dans la fonction publique, le Premier ministre puis vous-même avez au contraire confirmé cet objectif. est-ce une nouvelle traduction du « en même temps » ? C'est surtout en contradiction totale avec ce qu'exprime le pays, à savoir la nécessité de renforcer les équipes soignantes dans les hôpitaux, de réduire les effectifs dans les classes, de reconquérir l'égalité républicaine grâce à des services publics de proximité, modernisés, à même de faire reculer les inégalités. Je veux en premier lieu souligner les conséquences de votre projet en matière d'éducation. Nous connaissons une crise de recrutement dans le métier d'enseignant, ainsi qu'une augmentation très inquiétante du nombre de démissions, encore récemment relevée dans le bilan social de l'éducation nationale. redonner attractivité et reconnaissance à la profession. Vous choisissez une réponse court-termiste en généralisant le recours aux contractuels, alors que 20 % des agents de l'éducation nationale le sont déjà. Pour les seuls enseignants, le nombre a presque doublé en dix ans. Cela risque de se traduire par une dégradation de la qualité des enseignements. Car la contractualisation ne signifie pas seulement précarité et instabilité pour les agents. Elle signifie aussi moindre exigence du recrutement, manque de formation et d'expérience, et par conséquent moindre qualité de l'enseignement dispensé. À l'inverse exact du besoin de renforcement de la formation des enseignants, que nous avons identifié, au Sénat, à plusieurs reprises.

Prendre en compte les nouveaux besoins, comme celui d'accompagner les enfants en situation de handicap, dans le cadre d'une école inclusive, voilà qui contribuerait à une modernisation de la fonction publique ! Il est d'autant plus regrettable de ne pas s'engager dans cette voie qu'un consensus se dessine aujourd'hui autour de la nécessité de sécuriser et de professionnaliser ces personnels. Ainsi pourrait être créé un corps de la fonction publique, afin de répondre à un besoin qui constitue objectivement une mission de service public. Il pourrait s'agir de l'une des mesures phares d'une loi ayant pour ambition de moderniser la fonction publique, plutôt que de la démanteler. Je souhaite aussi évoquer les agents de la direction générale des finances publiques, qui font face à un plan social déguisé accompagnant la fermeture de nombreuses trésoreries dans nos territoires, alors même que la mission de service public de celles-ci est essentielle pour les particuliers, mais aussi pour les élus des petites communes qui ont besoin de ces services, de gérer les finances communales. Enfin, le transfert des conseillers techniques sportifs aux fédérations, adopté par l'Assemblée nationale, est une mesure particulièrement funeste,

Paris. La ministre des sports a indiqué qu'elle n'utiliserait pas cette disposition. Mais le plus sûr serait évidemment de la supprimer du texte. Vous pouvez compter sur nous pour intervenir en ce sens ! La parole

secrétaire d'État, vous nous annonciez la couleur en demandant à l'administration de faire sa « révolution culturelle ». Derrière ce vocabulaire empreint de sobriété, si caractéristique de la Macronie, que doit-on imaginer ? Plus de moyens, une meilleure écoute des demandes des agents, un renforcement de la fonction publique ? Parce qu'après tout cette fonction publique, qui est un atout pour notre pays, mérite bien cela, ne croyez-vous pas ? Les bons chiffres économiques dont vous vous félicitez régulièrement, les investissements étrangers de plus en plus nombreux, ne croyez-vous pas qu'ils sont dus aussi à l'avantage compétitif que représente le maillage du service public dans notre pays ? On aurait donc pu imaginer que vous renforceriez la fonction publique. Mais de renforcement, il n'y aura pas. Vous vous abritez derrière les totems de la souplesse, de l'agilité, des managers. Il est vrai qu'en termes de souplesse idéologique et de gestion des ressources humaines vertueuse M. Macron est un spécialiste. L'Élysée a pourtant fait l'expérience des risques liés au recrutement de contractuels aux fiches de poste mal libellées et au profil incertain Ces totems trompeurs dissimulent mal une orientation très libérale. Lors de la dernière campagne présidentielle, M. Fillon avait inquiété une partie des agents de l'État en évoquant 600 000 suppressions de postes dans la fonction publique.

Qu'importe, puisque vous allez mettre en place la boîte à outils pour fragiliser durablement la fonction publique. Vous faites du « Fillon light » : il y a moins de suppressions de postes, mais le goût de la fragilisation du service public est bien le même. Dans la période, le premier message à envoyer aux fonctionnaires, qu'ils travaillent aux urgences, dans les prisons, à l'école, sur les routes, consiste à les assurer de notre fierté, de nos encouragements et de notre écoute. À l'inverse, vous faites le choix de dépouiller les instances de dialogue social de leurs attributions. s'ouvre le procès de France Télécom, groupe qui incarne à merveille les différences entre une gestion de service public et un management libéral à l'anglo-saxonne, vous exposez les trois versants de la fonction publique à cette culture qui risque de précariser les agents publics et d'affaiblir le service public ! Quand la presse se fait l'écho de harcèlement envers des déléguées départementales aux droits des femmes, vous revoyez à la baisse les exigences des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, issues de l'accord du 30 novembre 2018 ! Votre projet de loi abandonne ainsi la trajectoire ambitieuse lancée sous le précédent quinquennat. De 2012 à 2017, l'objectif de primo-nomination féminine a été relevé de 20 % à 40 %. Une politique volontariste qui a fait la preuve de son efficacité, mais qui n'est, hélas, pas poursuivie. L'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat, ce ne sera pas pour la fonction publique.

Elles ne traiteront plus de mobilité, de mutation, d'avancement et de promotion. Comment ces femmes défendront-elles leurs droits demain, alors même qu'aujourd'hui elles doivent lutter quand des structures adéquates existent pourtant ? Je comprendrais, monsieur le secrétaire d'État, que vous n'appréciiez pas mon intervention. Mais j'aimerais que vous vous prononciez sur le cas de ces féministes fonctionnaires du quotidien. Je comprendrais aussi que mon argumentaire

Pour lutter contre la précarité, nous voulons élargir l'assiette de la prime de précarité à l'ensemble des CDD et limiter le nombre de renouvellements de CDD possible. Alors que vous ouvrez la porte à d'innombrables mouvements de personnel en partance de la fonction publique, nous souhaitons renforcer les obligations déontologiques

Pour pallier la perte d'attractivité induite par votre réforme, nous souhaitons ouvrir certains concours de la fonction publique territoriale aux candidats justifiant d'une certification professionnelle, et améliorer les possibilités de proroger les présences sur les listes d'aptitude. Concernant le recours accru au contrat, nous souhaitons étendre la règle selon laquelle un emploi public ne peut être réservé à un contractuel, mettre en place les mêmes conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle entre titulaires et contractuels, veiller à éviter les écarts de salaire entre eux. Nous proposons également un droit à la déconnexion pour les agents publics et souhaitons aligner la fonction publique sur le régime plus favorable du code du travail en matière de congés pour décès familiaux. Nous avons été stoppés par l'article 40 de la Constitution, mais nous invitons le Gouvernement à reprendre certaines de nos propositions à son compte. Autre proposition que nous avons déjà faite par le passé : nous voulons revenir sur le jour de carence pour les fonctionnaires. Mais cet amendement a, lui aussi, été retoqué sur le fondement de l'article 40 ... Les premiers résultats relativisent pourtant les bienfaits de cette mesure, que vous aurez l'occasion de nous présenter, monsieur le secrétaire J'aimerais sortir des propositions concrètes pour aborder un point qui me tient à coeur : la manière. Monsieur le président Bas, madame, monsieur les rapporteurs, j'ai personnellement trouvé exaspérantes les conditions d'examen de ce projet de loi en commission. On sait que le Gouvernement donne un sens très personnel au mot « concertation ». Ainsi, après quinze mois de concertation et alors que tous les syndicats sont hostiles à ce texte, on nous parle de nouveau contrat social. C'est, hélas, le lot quotidien des parlementaires ! Nous avons travaillé sur ce texte dans des conditions qui ne permettent pas d'être de bons managers, comme dirait M. Dussopt. Nous travaillons vite et mal. Nous avons passé à peine une matinée en commission sur ce projet de loi dont l'examen va nous réunir de nombreux jours et nuits en séance. La procédure accélérée rencontre ses limites Pendant ce temps, le Président de la République ne cesse de répéter que le Parlement ne travaille pas assez vite. On croit rêver ! Le groupe socialiste, vous l'aurez compris, tentera malgré tout de remplir son office en ayant en tête les surveillants de prison, les enseignants, les policiers, les délégués aux droits des femmes, les agents des lycées.

Aujourd'hui, elle emploie près de 5,5 millions d'agents, soit un ratio de 72 agents pour 1 000 habitants. À titre indicatif, la moyenne européenne est de 60 pour 1 000 habitants. Fruit d'une concertation lancée dès le printemps 2018, sujet fort du grand débat, le projet de loi de transformation de la fonction publique qui nous est présenté aujourd'hui entend « bâtir la fonction publique du XXI siècle avec plus de souplesse et de mobilité Il affiche donc, tout du moins dans son intitulé, une ambition certaine. Il vise à moderniser le statut de la fonction publique et les conditions de travail, à s'adapter aux réalités du terrain régulièrement décrites par les élus. À ce titre, ce texte prévoit un recours accru aux contractuels, une fusion des instances représentatives du personnel, encourage la rémunération au mérite et touche à l'harmonisation du temps de travail. Il entre dans une nouvelle logique, tournée vers une politique de management, que l'on peut retrouver dans d'autres pays européens tels que l'Allemagne ou le Portugal. Il s'agit donc avant tout d'un texte technique, dont on peut regretter qu'il ne donne pas une vision claire quant aux missions des agents publics, dans un contexte agité de refonte de notre architecture institutionnelle. Il a cependant le mérite de comporter des outils pratiques et concrets, que le Sénat a renforcés pour conférer les moyens d'agir aux employeurs publics. En sa qualité de chambre des territoires, le Sénat travaille depuis de nombreuses années sur ce sujet.

La commission des lois, guidée par l'excellent travail des rapporteurs, Catherine Di Folco et Loïc Hervé, a donc retravaillé le texte en profondeur et l'a enrichi de 154 amendements, autour de trois objectifs mieux répondre aux attentes des employeurs territoriaux ; mieux récompenser le mérite des agents ; mieux accompagner les agents handicapés. Ces trois axes illustrent à la fois le pragmatisme sénatorial, l'écoute de la Haute Assemblée, sa volonté forte d'intégrer et de faire en sorte que chacun trouve sa place dans la société. Les 50 000 employeurs territoriaux attendent des réponses et de la souplesse face aux défis et aux contraintes auxquels ils doivent faire face. Les contraintes sont connues depuis plusieurs années : ce sont les normes, les coupes budgétaires, les transferts de compétences sans moyens supplémentaires, ou encore des mesures qui ont fortement affecté les petites communes, comme la suppression des contrats aidés décidée à quelques jours de la rentrée scolaire de 2017. Les élus locaux employeurs ont besoin d'information et de visibilité : c'est en ce sens que le Sénat, par l'intermédiaire de la commission des lois, a introduit l'obligation de publier une feuille de route triennale dans laquelle l'État indiquerait l'incidence financière de ses décisions en matière de ressources humaines sur les budgets locaux. Cette obligation de visibilité et de projection devrait permettre aux collectivités de mieux gérer leur masse salariale, de mieux programmer les recrutements dans l'intérêt des agents et de la collectivité. Car le poids budgétaire des agents représente en moyenne, sachons-le, 35 % du budget des collectivités. La souplesse de la gestion des ressources humaines, quasi généralisée en Europe, est devenue une condition de performance et d'adaptation aux réalités locales. Il est donc important que les élus puissent assumer pleinement leur responsabilité d'employeur. Ils doivent pouvoir prendre appui pour cela sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs Dans le même temps, les règles présidant au recrutement, à l'évolution professionnelle, à la formation et au management des agents territoriaux doivent être assouplies. Ainsi, le projet de loi permet de recruter indifféremment un fonctionnaire ou un agent contractuel sur l'ensemble des emplois de direction de la fonction publique et dans les établissements publics de l'État. Les collectivités de moins de 1 000 habitants peuvent également recruter par voie de contrat sur l'ensemble de leurs emplois permanents. Le Sénat a souhaité aller plus loin en prévoyant l'élargissement de la possibilité du recours aux agents contractuels, l'encouragement au recrutement sur titres, ou encore plus spécifiquement la facilitation de l'intégration des policiers nationaux et des gendarmes dans la police municipale. Ces dispositions, que la Haute Assemblée avait déjà pu évoquer, devraient conférer à l'employeur une maîtrise dynamique de sa masse salariale, ce à quoi nous sommes tous attachés. Dans un deuxième temps, l'accent a été porté sur l'encouragement et la gestion de carrière des agents au travers de la rémunération au mérite. Celle-ci est la première attente des employeurs, comme le révèle une étude du Sénat. Véritable serpent de mer, elle fait peu à peu son nid.

Elle permet d'influer sur la motivation, donc sur la performance. Elle doit s'appuyer sur un entretien professionnel objectivé. Sur l'initiative des rapporteurs, les primes des agents prendront désormais en compte les résultats du service, et pas uniquement les résultats individuels. Fixer des objectifs collectifs peut en effet constituer un levier managérial efficace, notamment pour des missions d'exécution. De même, le régime indemnitaire pourra prendre en considération les spécificités territoriales, auxquelles le Sénat est particulièrement attaché, notamment pour encourager les agents publics à s'installer dans des zones enclavées. Le Sénat utilise ainsi les leviers pour lutter contre la désertification de nos territoires et le sentiment d'abandon qui s'y développe. Dans un troisième temps, le recours à l'apprentissage a été renforcé dans la fonction publique territoriale. L'apprentissage est un levier majeur pour la formation des jeunes, par la transmission du savoir-faire. C'est un sujet auquel je suis particulièrement attachée, puisqu'au coeur de l'action des missions locales. Il permet d'intégrer les jeunes les plus éloignés de la formation par une dimension pratique, tout en leur donnant une première expérience professionnelle au contact de la réalité du monde du travail. permet aussi de multiplier les chances du futur diplômé de trouver un emploi. Les apprentis apportent un regard neuf, une vision nouvelle dans la structure d'accueil, tout en contribuant dans la fonction publique notamment à diversifier les filières de recrutement. Les administrations publiques peuvent recourir à l'apprentissage depuis la loi du 17 juillet 1992. Pourtant, les collectivités, qui ne peuvent bénéficier des incitations financières prévues pour les entreprises, peinent à recruter des apprentis.

Enfin, la commission des lois a souhaité renforcer l'intégration des personnes en situation de handicap. Avec la loi de 1975, puis celle de 2005, a été engagée une politique inclusive de la personne en situation de handicap au coeur de la société. Aujourd'hui, sur un total de 938 000 travailleurs en situation de handicap, un peu plus de 250 000 sont des agents publics, soit 22 %. Un autre signe encourageant est la progression du taux d'emploi légal des personnes handicapées, qui est passé de 3,74 % en 2006 à 5,61 % en 2018.

Sera ainsi autorisée une expérimentation pour pérenniser le financement du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, actuellement en péril. Si le modèle économique de ce fonds repose sur une logique incitative, il subit actuellement un effet de ciseaux ciseaux : depuis 2013, ses dépenses d'intervention sont supérieures aux contributions reçues. Le nouveau modèle prévu s'organiserait autour d'une part fixe, soit 0,1 %, et d'une part variable basée sur le mécanisme du bonus-malus. Est également prévue l'intégration dans la fonction publique des apprentis en situation de handicap, sous réserve de leur aptitude professionnelle. Cette disposition permettra de renforcer l'accès à l'emploi public des personnes handicapées, tout en s'inscrivant En outre, un droit à la portabilité des aménagements de poste, pour que les agents puissent conserver leur aménagement lorsqu'ils changent d'employeur, a été entériné. Là encore, cette proposition relève d'une vision pragmatique et efficace. et efficace. Le texte qui nous est soumis a été substantiellement enrichi par la commission des lois. Il permettra de doter les employeurs d'outils rendant possible une gestion stratégique de la masse salariale, et ce dans une perspective d'évolution de la répartition des compétences et des métiers de la fonction publique. Les volets de l'accès à la fonction publique par la voie de l'apprentissage et du renforcement de l'intégration des personnes handicapées viennent compléter ce dispositif,

On peut dire que votre texte affiche une ambition qui n'est pas mince ! Transformer la fonction publique, cela signifie faire évoluer les situations, les pratiques et le quotidien de près de 5,5 millions d'agents publics en France. Cela implique aussi d'améliorer le recrutement, la formation et le déroulement des carrières. Cela signifie, enfin, se pencher sur les principes déontologiques qui organisent la fonction publique. En somme, il s'agirait de réinventer celle-ci sans revenir sur la tradition française du service public sur les grandes lois statutaires de 1983 et 1984. Vous affirmez que votre projet de loi parvient à cet équilibre, qu'il transforme la fonction publique sans en renier les fondements, voire même qu'il « refonde le contrat social » qui lie les agents au service de notre pays. Qu'en est-il de la réalité de ces dires ? Devant le bric-à-brac de mesures contenues dans le présent texte, on cherche en vain une vision d'ensemble. Le président de la commission des lois, Philippe Bas, avec le sens de la formule et de la litote qui lui est propre, évoquait une « boîte à outils » ! Cette métaphore traduit le caractère désordonné et parfois hétéroclite du projet Sans prétendre à l'exhaustivité, je reviendrai sur quelques-unes de ces mesures. En premier lieu, il me semble qu'un certain nombre de dispositions répondent aux attentes des employeurs territoriaux et vont dans le bon sens.

Comme il faut être bienveillant-et nous le sommes -, je préfère saluer votre souplesse et votre agilité, qui ne sont pas anecdotiques, ainsi que la vivacité avec laquelle vous défendez une telle disposition. Disons que cela relève des mystères de la conversion ! L'engagement politique comporte sa part d'énigme, il faut le reconnaître. Cela confirme au moins que ce sont souvent les plus fraîchement convertis à une cause nouvelle qui se révèlent parfois les plus fervents et les plus ardents pour la défendre. la défendre. Je retiens également un intéressement croissant des fonctionnaires à l'activité de leur service, qui me semble constituer une évolution positive, au même titre que l'harmonisation du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, j'espère que la fusion de la HATVP et de la commission de déontologie de la fonction publique, fruit des travaux de l'Assemblée nationale, pourra favoriser la diffusion, toujours plus large, d'une culture de la déontologie dans la fonction publique. Enfin, le projet de loi comporte des mesures intéressantes relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qu'il nous faut saluer, ainsi que des mesures en faveur des personnes handicapées.

Je souhaite que ces éléments trouvent leur place dans le texte final. Réformer la fonction publique est utile et même nécessaire. J'espère que la discussion de ce projet de loi fera émerger des voies et des outils concrets pour cela. Car il faut que ce texte améliore très concrètement la qualité des services rendus par les administrations aux Français, en particulier dans les territoires, tout en offrant aux agents publics une plus grande fluidité de leurs parcours. Cela étant dit, sans céder au pessimisme, je n'attends pas de ce texte le changement profond que nos concitoyens souhaitent. Un certain nombre de questions demeurent en effet. Par exemple, quelles missions doivent être remplies par des fonctionnaires, et quelles missions peuvent l'être par des agents contractuels ? Recourir de manière accrue aux contractuels peut certainement présenter un intérêt. Mais le faire sans l'inscrire dans une démarche plus cohérente revient à prendre le risque du désordre dans les services et de l'incertitude sur la maîtrise des masses financières en jeu. Une telle démarche impliquerait aussi un travail plus approfondi sur les modalités de recrutement et des concours. Or le projet de loi n'offre pas de réflexion globale satisfaisante sur ces sujets cruciaux. On n'y retrouve guère les ambitions d'une réforme politique d'ampleur. Au lieu de cela, ce texte privilégie un chapelet de mesures techniques qui ne sont parfois pas sans contradiction entre elles. Cette situation laisse craindre une occasion manquée, même après quinze mois de discussions entre le Gouvernement et les représentants des agents publics.

Sur un sujet aussi important que celui de l'avenir de la fonction publique, il serait préférable de se borner à recourir aux ordonnances dans les cas spécifiques où leur plus-value paraît incontestable. Par exemple, on ne peut qu'accueillir favorablement la codification, par ordonnance et à droit constant, du droit de la fonction publique. On pourra toujours considérer que ce projet de loi a le mérite de mettre le sujet de la fonction publique sur la table, et, conformément à ses habitudes, le Sénat s'efforcera d'apporter une contribution riche et utile.

Ceux-ci ont fait oeuvre d'orfèvre, afin d'améliorer le texte qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale. Leur attention s'est notamment portée vers les enjeux locaux, comme les conditions de la mobilité des personnels vers les polices municipales. Nous restons donc sur notre faim, même si nous nous efforcerons d'être une force de proposition agissant en faveur d'une réforme réelle de la fonction publique, afin de pouvoir aboutir à un texte qui soit véritablement une amélioration.

la question à la fois de la place, du rôle et de l'ampleur du recrutement des contractuels. Un certain nombre de dispositions adoptées par votre commission des lois peuvent paraître, en l'état des expressions des associations d'élus, contradictoires avec les attentes de ces derniers, notamment sur la fonction publique territoriale. Nous devrons aussi revenir, au-delà de la question de l'ampleur de l'ouverture des recrutements contractuels, sur le rôle de ceux-ci.

et bénéficient des mêmes droits que les agents titulaires, garantissant ainsi leur indépendance et leur plein rattachement, si vous me permettez cette expression, au statut. Nous devrons aussi débattre du dialogue social et du rôle des commissions administratives paritaires,

du format et de la nature même des épreuves ou des matières soumises à concours. L'ensemble des questions relatives aux concours relève du champ réglementaire : c'est la raison pour laquelle nous n'avons introduit aucune disposition dans le texte de loi. Mais les travaux sont en cours ; nous en sommes à la deuxième ou troisième réunion de travail

la volonté du Gouvernement, exprimée par le Président de la République et par le Premier ministre, à la fois d'identifier les services pouvant être exercés, parce que ce sont des services d'instruction, dans des territoires ruraux ou périurbains, et de rappeler, comme il le fait depuis 2018, et encore récemment par la circulaire du 12 juin dernier,

un tropisme qui a toujours conduit à supprimer des postes plutôt dans les services déconcentrés que dans les administrations centrales, il est nécessaire de mener une véritable entreprise de déconcentration et d'accompagner les mouvements fonctionnels et géographiques des agents. Le texte que je présente devant vous permettra de faire cet accompagnement dans de bonnes conditions, et pour ces et pour les services. grande ouverture d'esprit dont vous avez témoigné dans votre réponse à mes collègues qui se sont exprimés à la tribune. Je veux souligner que la matérialisation de cette ouverture d'esprit, de mon point de vue de président de la commission des lois, et mes collègues auront certainement leur propre opinion en l'espèce, devrait porter sur un certain nombre de points du texte tel que nous avons essayé de le retravailler. Nous avons abordé l'examen de ce projet de loi avec un préjugé qui n'était pas défavorable. Mais certains sujets nous tiennent à coeur, et je vais les citer en vrac, pour que vous soyez bien averti de ce qui est important pour nous : l'apprentissage, notamment dans les collectivités locales, de nouvelles souplesses de gestion pour les exécutifs locaux, la fin d'un certain nombre d'abus qui n'ont pas été corrigés corrigés par les gouvernements successifs, notamment s'agissant des personnes momentanément privées d'emploi- mais il y a d'autres exemples -, et plus important pour l'insertion des personnes handicapées- sur ce point, je veux de nouveau saluer le travail qui a été fait par Catherine Di Folco et André Marie ici présent. Didier Marie !

de loi de transformation de la fonction publique qui vise à moderniser le statut et les conditions de travail dans la fonction publique, en assouplissant les modalités de recrutement des agents publics. En effet, il s'agit là de la réponse du Gouvernement à la dégradation des services publics. Les services publics d'aujourd'hui sont-ils en adéquation avec les besoins des usagers ? Non Faut-il redonner toute leur place aux services publics dans toute leur diversité ? Bien entendu ! Ce projet de loi est-il la réponse adaptée ? Je n'en suis pas sûr ! Je tiens à rappeler à cette assemblée le rapport annuel sans concession du Défenseur des droits, Jacques Toubon, qui insiste sur l'explosion des inégalités, de la précarité, de la pauvreté. Il dénonce principalement la réduction du périmètre des services publics, fruit de la privatisation des services organisés en réseau- la poste, les télécommunications, l'eau, le gaz, etc. ; le désengagement de l'État de ses obligations, par le recours à la délégation massive de certains services publics ; les restrictions budgétaires frappant les services publics demeurés dans le giron de l'État. D'ailleurs, les chiffres sont éloquents : plus de 140 000 demandes d'interventions ou de conseils auprès du Défenseur des droits, 95 000 dossiers de réclamations, dont 55 785 concernant les relations avec les services publics,

Mais le texte qui nous est proposé sera, en l'état, générateur d'insécurité juridique en raison du manque de précisions sur certaines notions et certains dispositifs, notamment le contrat de projet. De la même manière, que se passera-t-il si un fonctionnaire refuse un détachement ? La parole Marie, sur l'article. Le dialogue social peut se définir comme l'ensemble des processus d'échanges organisés entre représentants des employeurs et des salariés. Cette définition s'applique aussi bien au secteur privé qu'au secteur public. Mais les spécificités de la fonction publique singularisent largement le dialogue social qui s'exerce en son sein, les fonctionnaires étant soumis à un régime juridique exorbitant du droit commun. La conception française du rôle de l'État dans la société a déterminé le mode de régulation des rapports de celui-ci avec ses agents. La place reconnue à la puissance publique dans la définition de l'intérêt général justifie la prédominance du principe hiérarchique dans son organisation, et donc la situation statutaire des fonctionnaires. C'est l'État employeur qui fixe unilatéralement les conditions d'emploi de ses agents, ainsi que l'étendue de leurs droits et de leurs obligations. Ce dialogue social dans la fonction publique doit ainsi emprunter un chemin de crête entre principe hiérarchique et participation. En 1946, le dialogue social fut conçu comme un compromis visant à contrebalancer la rigidité de la subordination statutaire par une consécration des garanties individuelles et collectives des fonctionnaires. Ce principe de participation veut que les agents soient associés aux mesures qui les concernent, qu'elles soient individuelles ou collectives. C'est l'application à la fonction publique du principe posé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

C'est ce principe de participation, qui a pourtant été réaffirmé comme principe général du droit par le Conseil constitutionnel en juillet 1977, que l'article 1 du présent projet de loi attaque en réduisant la capacité d'intervention des délégués du personnel, en les privant notamment, par le dessaisissement des CAP, de l'examen des situations individuelles et en réduisant leur champ d'action dans le domaine de la prévention de la santé des agents par la fusion des comités techniques et des CHSCT. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons les amendements de suppression de cet article.

effet, sous couvert de réaffirmer le principe constitutionnel de participation des agents publics, notamment par l'intermédiaire de leurs délégués, au fonctionnement des services publics, l'article 1 vise en réalité à supprimer la mention conférant aux syndicats des décisions individuelles relatives aux carrières des fonctionnaires. Le mécanisme est habile, puisque cet article renvoie à un décret la définition des décisions individuelles qui relèvent de ce principe de participation, remplaçant ce dernier par un principe général de participation à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines, ce qui est- vous me l'accorderez -totalement différent. Je vous rappelle, mes chers collègues, que le principe de participation est né après-guerre, inspiration ayant été prise notamment des travaux du Conseil national de la Résistance participant à reconnaître des droits économiques et sociaux collectifs, qu'il constitue l'un des piliers de notre démocratie comme principe général du droit, reconnu comme tel en 1977. Dans la lignée idéologique de l'ensemble du projet de loi, le dispositif proposé réduit néanmoins de manière significative la démocratie sociale au sein de la fonction publique, en amenuisant de fait le rôle des commissions administratives paritaires, même si la commission des lois a rétabli ces commissions dans certaines de leurs prérogatives. Cette décision est tout à fait symptomatique de la volonté du Gouvernement de transformer cette instance paritaire en lieu de consultation purement formelle et d'en limiter le nombre. Le dessein au fond est bien celui-là, tel qu'exposé dans l'étude d'impact, puisqu'il est indiqué que la réforme des CAP devrait se traduire par une incidence budgétaire positive. Cette disposition va donc dans le sens de l'austérité budgétaire réalisée sur le dos de la démocratie sociale. administratives paritaires sont pourtant essentielles à la vitalité du dialogue social au sein de la fonction publique. Elles constituent un rempart contre les intérêts particuliers contre l'arbitraire auquel peuvent être soumis un certain nombre de fonctionnaires. Nous demandons donc la suppression de l'article 1, afin que les syndicats puissent continuer d'influer sur les décisions relatives aux carrières des fonctionnaires, et ainsi concourir au bon fonctionnement des services publics. La parole

permet la fusion des instances du dialogue social et puise directement son inspiration dans les dispositions qui ont été appliquées aux entreprises privées, il y a un peu plus de dix-huit mois. Je tiens à faire le parallèle et à vous alerter, mes chers collègues, sur ce point. Le constat des organisations syndicales, que nous avons consultées pour faire le point sur les dispositions en vigueur depuis leur adoption il y a dix-huit mois, est unanime. Quand nous leur demandons si la fusion des instances a été de nature à renforcer le dialogue social, elles répondent sans équivoque que tel n'est pas le cas, que les accords conclus sont de piètre qualité, et que, si les entreprises qui bénéficiaient d'un dialogue social de bonne qualité l'ont conservé, on se contente, pour le reste, du minimum légal. Je crains que l'erreur qui a été commise à l'égard du secteur privé ne finisse par contaminer la fonction publique, dont la réforme s'inspire de cette fusion des instances du dialogue social. Je le dis en particulier s'agissant de la suppression des CHSCT, parce que je redoute que la question de la sécurité et de la santé au travail ne finisse par devenir secondaire dans la discussion menée par un certain nombre des partenaires sociaux au sein de ces instances regroupées. Je suis d'ailleurs intéressé de connaître la position de M. le secrétaire d'État, qui, me semble-t-il, a changé d'avis en quelque temps sur ce sujet. De plus, avec cet article, on court le risque de réduire les commissions administratives paritaires à peu de chose, alors qu'elles étaient auparavant consultées sur les situations individuelles sans toutefois disposer de pouvoir de décision. étaient, en revanche, un facteur de transparence, un moyen d'éviter que l'arbitraire ne s'immisce dans l'avancement des agents- je mets ce risque de favoritisme en regard de l'usage inconsidéré que vous voulez faire du contrat en concurrence avec le statut et, surtout, avec le concours, Chaque fois que vous affaiblissez les protections statutaires, vous affaiblissez non pas tant la protection des agents que celle de l'ordre public et de l'intérêt général que ceux-ci défendent. Vous mettez en danger la défense de cet intérêt général par les fonctionnaires, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cet article soit supprimé.

Le projet de loi issu des travaux de la commission des lois ne reprend pas l'ensemble des modifications relatives aux organes paritaires des trois versants de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les compétences des CAP, comme Mme Cukierman l'a elle-même Néanmoins, les options que nous avons retenues rendent nécessaire la modification prévue à l'article 1, en particulier en ce qui concerne la mention des décisions individuelles. L'avis de

Par ailleurs, nous prévoyons qu'à partir de 300 équivalents temps plein dans la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière et de 200, à la demande de l'AMF particulièrement, dans la fonction publique territoriale une formation spécialisée soit chargée de traiter les questions d'hygiène et de sécurité, ce qui devrait rassurer M. Marie.

permettra, de surcroît, de simplifier les conditions du dialogue social entre les administrations et les représentants des agents, s'agissant par exemple des évolutions futures de l'organisation du travail induites par les nouvelles technologies. » Enfin, j'ajoute que nous avons prévu que cette nouvelle instance couvre l'ensemble des compétences des comités techniques et des CHSCT et que lui soit ajoutée une compétence nouvelle : la définition des lignes directrices de gestion des ressources humaines, les sujets concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou encore les règles d'accès à la mobilité et à la formation.

mon sens, il s'agit d'un affaiblissement très important du dialogue social qui est à la fois néfaste bien évidemment pour les agents, mais aussi pour les employeurs, car, dans le cadre du dialogue social actuel, les échanges permettaient également de les

la déontologie des fonctionnaires relève de la seule compétence du législateur pour ce qui est de fixer les règles applicables, et de l'autorité de l'administration et de la HATVP, pour en apprécier l'application. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut,

Nous souhaitons supprimer la disposition qui indique qu'à l'avenir un décret établira une liste des décisions individuelles sur lesquelles les CAP se concentreront, et donc en creux toutes les décisions qui ne relèveront plus de ces instances. Il s'agit en réalité de réduire le périmètre du principe de participation des agents. Nous tenons alors à vous alerter. Que va-t-il se produire en l'absence de consultation des commissions administratives paritaires ? Le doute va s'installer sur l'arbitraire de la décision, qui a souvent de lourds impacts personnels. Nous pouvons craindre une augmentation du contentieux, et par conséquent de la conflictualité au sein de l'administration. En fait, une telle réforme aboutira à une moins bonne prise en compte des situations individuelles et collectives, à un manque de transparence et à un accroissement des tensions au sein des administrations. Est-ce réellement cela la modernisation des instances de dialogue social ? Nous ne le croyons pas, particulièrement dans un contexte social déjà extrêmement compliqué. D'ailleurs, les syndicats représentatifs se sont unanimement opposés à cette disposition qui remet en cause non seulement le principe de participation, mais également leur utilité au bénéfice de ces mêmes agents. vous demandons donc de renoncer à ces économies d'échelle, comme vous dites, monsieur le secrétaire d'État, qui sont en réalité des économies de pacotille, et de conserver les instances de dialogue social, qui ont fait leurs preuves par leur composition paritaire pour traduire les principes fondateurs de la fonction publique de responsabilité et d'impartialité. Nous demandons par cet amendement la suppression du renvoi au décret pour la définition des décisions individuelles qui ne relèveraient plus du principe de participation. Quel

retenues par la commission des lois. Au-delà, nous avons prévu dans le modèle d'organisation du dialogue social que nous proposons à la fois de la publicité, en particulier celle des barèmes, une délibération sur les lignes directrices de gestion,

de la fonction publique comme contrepartie de la liberté d'expression dont ces derniers bénéficient. Ce devoir de réserve implique que, lorsqu'ils s'expriment, les agents ne doivent pas adopter de position de nature à donner une image négative, discréditant leur administration ou leur hiérarchie. Pourtant, ce principe est d'origine prétorienne et demeure encore extra-statutaire, en dépit d'une tentative sénatoriale pour l'intégrer dans la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

et en mettant celle-ci directement en relation avec les fonctions et la situation de l'agent. Cette formulation reprend en partie les termes de la décision fondatrice

avec tact et discernement. Cette jurisprudence est ancienne et bien ancrée. Le Conseil d'État a reconnu, dès 1935, qu'un agent de la chefferie du génie de Tunis pouvait être sanctionné pour avoir tenu des propos critiques envers le Gouvernement. L'amendement présente en outre plusieurs garanties : le devoir de réserve s'applique dans l'exercice de l'emploi, selon les fonctions exercées et la situation de l'agent. Ainsi, il comprend une exigence de proportionnalité et ne remet pas en cause la liberté d'expression du fonctionnaire citoyen.

À ce stade, il ne nous paraît toujours pas opportun de consacrer dans la loi le devoir de réserve. Pour nous- mais cela a également été rappelé -, celui-ci est d'abord et avant tout une construction jurisprudentielle, imposant aux fonctionnaires de faire preuve de modération dans l'expression de leurs opinions, dans l'exercice de leurs fonctions ou dans leur vie privée. Sa portée est variable. Il est apprécié, au cas par cas, en fonction de la nature des responsabilités de l'agent, de son rang, de sa catégorie hiérarchique, des circonstances, du ton et du cadre dans lesquels sont tenus les propos incriminés et nous savons, par exemple, que l'obligation est atténuée pour les responsables syndicaux. De plus, ce devoir découle déjà d'autres obligations consacrées dans la loi : la discrétion et le secret professionnel, ainsi que le devoir de neutralité et le respect du principe de laïcité. Parce que ces obligations figurent dans la loi

que de réduire leur liberté d'opinion et d'expression. Nous voterons contre cet amendement.

: La parole est à M. Jean-Claude Tissot. Le Gouvernement s'enorgueillit de l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. Ce n'est pas la première fois que nous occupons cette deuxième place, voire la première en Europe. notre pays repose sur nos infrastructures et sur la qualité de nos services publics de santé, d'éducation, d'administration, de justice, notamment sur l'intégrité et l'objectivité des fonctionnaires qui les servent. Les Français sont attachés à des services au-dessus de tout soupçon de partialité ou de conflit d'intérêts. Si le statut des fonctionnaires garantit la capacité de chacun d'entre eux de résister aux pressions, il n'en est pas de même des contractuels, sur lesquels peut peser la menace d'un non-renouvellement de contrat ou d'un refus de passage en CDI en cas de réticence à se soumettre à des pressions intéressées.

cet amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur. Les principes déontologiques et les mécanismes de lutte contre la corruption s'appliquent aux agents contractuels. Ces derniers ont également accès à un référent déontologue, qui peut répondre à leurs questions les plus concrètes. L'adoption de cet amendement pourrait même avoir un effet contraire, sans doute non souhaité par ses auteurs. Ces dispositions signifient-elles que les fonctionnaires ne bénéficient pas de ces garanties d'impartialité ? Il paraît donc plus sage d'en rester au droit en vigueur, qui apporte les garanties nécessaires. L'avis de la commission est défavorable.

modifier l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, pour y ajouter des dispositions non normatives à visée évocatoire. Cet article 25 est important. Il prévoit notamment que le fonctionnaire « exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » ; que « dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité » ; qu'il « exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité » et « à ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses » ; qu'il « traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. » L'article 25 sert donc de base légale aux sanctions pouvant être prononcées contre les fonctionnaires. Les deux rapporteurs ont, à juste titre, proposé la suppression des modifications adoptées par les députés,

aux agents contractuels du secteur public, en cohérence avec l'importance croissante de ceux-ci au sein de l'administration et l'intention du Gouvernement de renforcer leur proportion par le biais de ce projet de loi. Les agents contractuels représentent désormais 20 % des agents publics, mais pâtissent encore d'une faible protection législative, comme on le verra dans la suite

supérieurs, dès lors que ceux-ci présentent un lien avec les dispositions communes. Dans ce cas, et c'est ce qui nous contrarie, l'avis du Conseil commun se substituerait à celui du conseil supérieur du versant concerné. Nous aurions préféré que deux avis puissent coexister, instituant ainsi des complémentarités utiles. Mais non ! On choisit d'utiliser le Conseil commun pour museler les conseils supérieurs

consultation de l'administration de rattachement des personnels concernés. Chaque conseil supérieur doit être consulté sur tous les projets de texte ou de rapport intéressant la situation des agents de chaque versant de la fonction publique. Les conseils supérieurs, qui comptent chacun des représentants et des représentantes des employeurs et des personnels de chaque fonction publique, sont des instances d'expertise

de la commission ? Cet amendement tend à supprimer l'article 2 dans sa totalité. Comme vous, madame Apourceau-Poly, nous avons craint que les dispositions du projet de loi ne conduisent à un accroissement excessif des compétences du Conseil commun de la fonction publique au détriment des conseils supérieurs.

solution de compromis, subordonnant l'extension de compétence du Conseil commun à l'accord des présidents des conseils supérieurs de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

au motif qu'il risquait de placer les présidents des conseils supérieurs de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans une situation compliquée vis-à-vis des autres membres, nuisant ainsi au bon déroulement du dialogue social au sein de leurs instances.

Dans le même esprit que l'amendement précédent, nous demandons la suppression de la faculté donnée au Conseil commun de la fonction publique de se substituer à l'un des conseils supérieurs des trois versants de la fonction publique, qui connaissent des réalités très différentes. Pour ne prendre qu'un exemple, nous ne souhaitons pas que cette disposition permette au Gouvernement de court-circuiter le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et ce même avec l'accord de son président. Il ne nous paraît pas opportun que les projets de loi et d'acte réglementaire relevant de la fonction publique territoriale, intéressant les employeurs et les fonctionnaires territoriaux, fassent l'objet d'une délibération au sein d'une instance où ils seront beaucoup moins bien représentés, voire totalement minoritaires, en ce qui concerne les employés en tout cas. Le même raisonnement vaut évidemment pour les autres conseils supérieurs. Que le Conseil commun puisse se saisir et formuler un avis est une bonne chose ! Mais que cet avis supplante celui du conseil le plus concerné, où les acteurs sont le mieux représentés, n'en est pas une ! C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition.

Or, en 2015, seuls 8,5 % des agents se trouvaient en situation de mobilité : 4,5 % ont changé d'employeur public ; 4,2 % de zone d'emploi et 2,9 % de statut ou de situation d'emploi. Les primes et les différences de régimes indemnitaires constituent un frein aux souhaits de mobilité des agents, comme le soulignait déjà Jean-Ludovic Silicani dans son rapport publié en 2008 en 2008 : « malgré une politique active de fusion de corps, d'harmonisation statutaire et d'élargissement des viviers amorcée depuis plus d'une dizaine d'années et accélérée sur la période la plus récente, le corps reste, dans le système actuel, l'élément qui détermine ce que l'administration peut faire en termes de rémunération, de promotion et Ainsi, celle-ci ne peut pas offrir le même niveau de prime et les mêmes possibilités de promotion pour des agents n'appartement pas au même corps ou au même grade, mais assumant pourtant les mêmes fonctions. Outre qu'elle est manifestement inéquitable, cette situation est contre-productive ». Bien que des efforts de convergence aient été déployés au cours des dernières années, il semble que ces différences indemnitaires constituent toujours un frein à la mobilité des agents. Afin de s'emparer plus vigoureusement du problème, le présent amendement vise à donner compétence au Conseil commun de la fonction publique, l'instance consultative du dialogue syndical rassemblant toutes les fonctions publiques, pour travailler à la convergence des rémunérations entre les fonctions publiques. Cette convergence, est-il précisé, s'établirait à un niveau de responsabilité et de risque physique équivalent. Concrètement, il est proposé de confier à l'instance le suivi des évolutions des rémunérations dans toutes les fonctions publiques et la mission de formalisation des propositions annuelles en ce sens, à destination des pouvoirs législatif et réglementaire.

ses compétences actuelles lui permettent d'examiner toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques, notamment sur des thèmes tels que les évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique, la mobilité, les parcours professionnels, la formation professionnelle tout au long de la vie. Dès lors, madame Delattre,

comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes insuffisamment informés des avis, des analyses et des propositions des représentants du personnel.

l'amendement que nous présentons tend à ce que les procès-verbaux du Conseil commun et des conseils supérieurs soient communiqués au Parlement, avec l'étude d'impact, lorsqu'ils concernent des textes de portée législative relatifs à la fonction publique. Il y va de la bonne information des parlementaires et donc de la qualité de la loi. lorsque ces conseils sont consultés sur un projet de loi ou d'ordonnance. Pourquoi pas ? La commission émet un avis de sagesse

du secteur ... Or l'avis et les propositions des membres des instances sont publiés sur le site internet de l'administration concernée et peuvent d'ores et déjà être consultés à tout moment. En revanche, il nous paraît matériellement difficile d'annexer les procès-verbaux à l'exposé

1946 et reconnu principe général du droit par le Conseil constitutionnel, en 1977. Pour autant, la rédaction actuelle de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que le Conseil supérieur comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, sans référence aux agents contractuels. Dans la continuité de notre volonté d'assurer une protection sociale des agents contractuels publics équivalente à celle des fonctionnaires, nous souhaiterions adapter la composition du CSFPE au phénomène croissant de recours aux contractuels. En effet, comme le montrent les irrecevabilités financières soulevées à l'encontre de notre amendement visant à faire converger, à fonctions et compétences égales, les rémunérations des agents titulaires

En outre, on constate également l'importance du phénomène de recours abusif à des CDD, sans que le Conseil d'État juge bon de prononcer des requalifications lorsqu'il constate ces pratiques.

lors de l'interruption de la relation d'emploi en l'évaluant en fonction des avantages financiers auxquels l'agent contractuel aurait pu prétendre en cas de licenciement, s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, il s'agissait d'un agent d'entretien ayant été recruté pour les mêmes tâches, selon vingt-huit contrats et avenants successifs. Sur la base de ces constatations, il serait donc utile de prévoir, à tout le moins, que ces agents contractuels puissent être représentés au sein du CSFPE, au même titre que les agents titulaires, afin que le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion

des agents de la fonction publique territoriale avait institué le Centre national de formation de la fonction publique territoriale, le CNFFPT. Cet établissement public administratif était notamment chargé de la collecte des contributions financières des employeurs, ainsi que de la définition et de la mise en oeuvre des actions de formation en direction des agents de la fonction publique territoriale. Il était dirigé par un conseil d'administration, lequel gérait- à l'instar de ce qui prévaut dans le secteur privé privé -de manière paritaire les fonds de formation en associant des représentants des employeurs et des représentants des organisations syndicales représentatives dans la fonction publique territoriale. Or cet établissement public administratif a été supprimé et ses missions transférées au CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, par la loi du 13 De fait, ce texte a abrogé la gestion paritaire de la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale. Ce paritarisme a été rétabli

à la formation professionnelle. Cet amendement tend à revenir aux dispositions qui prévalaient avant la loi Hoeffel, afin d'accorder une plus grande place à la démocratie sociale et de rétablir le paritarisme comme principe de fonctionnement de l'ensemble des instances sur l'ensemble des délibérations.

et non ceux des syndicats, participent au scrutin lorsque les délibérations portent sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire, ainsi que sur le budget du CNFPT. Les collectivités territoriales étant les seules contributrices au budget du CNFPT, il nous semble normal qu'elles conservent la maîtrise du financement de cet organisme et qu'elles restent le garant de son équilibre.

la commission des lois impose au Gouvernement de présenter devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route triennale comportant les engagements, les objectifs en matière de gestion des ressources humaines et leurs conséquences pour les collectivités.

Il s'agit d'accroître la visibilité pour les élus locaux et de renforcer le dialogue. La fonction publique territoriale est trop souvent à la remorque des décisions de l'État, que ce soit sur la valeur du point d'indice ou sur les accords statutaires. L'accord Parcours professionnels, carrières et rémunérations coûte, par exemple, 770 millions d'euros aux collectivités territoriales, sans aucune compensation de l'État. J'imagine que Philippe Mouiller

symbolique. Nous viendrait-il à l'idée, en tant que sénateurs représentant les collectivités, d'inscrire dans la loi qu'il appartient à l'État de remettre au Conseil supérieur de la fonction publique ce qu'il préconise de manière pluriannuelle en matière de gestion des ressources humaines de nos collectivités,

et de mesurer l'intérêt de cette feuille de route triennale, laquelle permettrait d'éclairer les collectivités territoriales sur les orientations en matière de gestion des ressources humaines. Il va de soi que les